Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande que l'examen des deux conventions internationales examinées en procédure simplifiée, initialement inscrites à l'ordre du jour du jeudi 23 mai, soit avancé au mercredi 22 mai après-midi. Par ailleurs, le Sénat ne siégerait jeudi 23 mai qu'à titre éventuel pour la suite de l'examen du projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse. Acte est donné de cette demande.

notamment au titre de la contribution à l'aménagement du territoire. En effet, on le sait, les commerces physiques sont les principaux contributeurs à l'aménagement du territoire au travers de la fiscalité variée à laquelle ils peuvent être soumis. Le présent amendement tend à ce que leur assujettissement à la taxe des soit soumis à la condition de réalisation d'au moins 50 % de leur chiffre d'affaires au titre de ladite livraison de biens. Ce seuil vise à intégrer ces dernières dans le champ de l'application de la taxe tout en exonérant les acteurs présents dans le commerce physique et qui contribuent,

adoptée l'Insee. Prendre comme assiette les seuls services taxables n'est pas adapté au fonctionnement des firmes du secteur du numérique, dont les activités sont souvent transsectorielles. Dans ce cadre, se référer à la notion d'activité des plateformes telles que les réseaux internet, mobiles et de capteurs, y compris le commerce électronique, nous paraît mieux répondre aux enjeux qui sous-tendent la discussion de ce texte. L'amendement

et nous souhaiterions que vous vous y intéressiez sérieusement. De principe, car nous voulons répondre à une difficulté que beaucoup ont pointée ici l'inefficacité de notre système fiscal, qui, au regard du sujet qui nous occupe ce soir, est uniquement fondé sur l'établissement. Pour les géants du numérique, de telles fondations sont inopérantes. inopérantes. Reconnaître un établissement stable virtuel, basé sur une présence numérique considérée comme significative, est possible. Nous proposons des seuils clairs : une fourniture de services numériques à des utilisateurs supérieure à 7 000 000 euros

Cet amendement soulève certes une question de principe, mais il se veut aussi pragmatique : des États à la culture numérique importante ont intégré à leur système fiscal la notion d'établissement stable virtuel. Je citerai deux exemples, que vous devez connaître, monsieur le ministre : l'Inde et Israël. La Commission européenne elle-même utilise dans son paquet sur la fiscalité numérique de novembre 2018 la notion de présence significative.

L'article 1 définit comme redevables de la taxe sur les services numériques les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 750 millions d'euros au niveau mondial et 25 millions d'euros en France. Cette taxe devrait s'appliquer dès 2019, donc sur le chiffre d'affaires réalisé en 2018. Cela ne tient pas compte- et cet amendement est du même esprit que les précédents -d'une caractéristique importante du secteur, à savoir la présence de sociétés jeunes est en forte croissance. croissance. Par ailleurs, comme la taxe est assise sur le chiffre d'affaires, elle s'appliquerait donc aussi aux sociétés réalisant peu ou pas de bénéfices, ce qui représente à l'évidence un risque pour leur pérennité. Le double critère de 750 millions et de 25 millions d'euros crée un effet de seuil potentiellement dommageable aux start-up en particulier. C'est pourquoi nous proposons d'atténuer cet effet en considérant comme redevables de la TSN les sociétés dont le chiffre d'affaires aurait dépassé ces seuils au minimum au cours des trois années consécutives, ce qui permettrait à la fois de préserver leur croissance et de leur donner le temps d'accéder à une certaine profitabilité. Bien sûr, cette modification ne bénéficierait pas aux gros acteurs, qui dépassent déjà de longue date ces seuils. C'est la même logique qui

Cela crée une différence de traitement forte entre les acteurs du secteur, qui ne nous apparaît pas opportune et qui pourrait même se révéler contre-productive. Le présent amendement vise donc à abaisser d'environ 40 % le seuil national en question.

rappeler que nous avons travaillé pendant près de deux ans sur les contours de cette taxe avec les services juridiques et fiscaux de la Commission européenne. Nous avons trouvé un équilibre autour d'un chiffre d'affaires mondial de 750 millions d'euros et d'un chiffre d'affaires national de 25 millions d'euros. Nous avons trouvé un équilibre autour de la base fiscale,

Je voudrais profiter de ce débat pour répondre à certaines questions et lever certaines ambiguïtés. La taxe porte sur trois catégories de services taxables,

Ces trois catégories concernent l'intermédiation entre internautes avec les plateformes, la fourniture de prestations de ciblage publicitaire, ce qui vous permet de recevoir toutes les secondes sur vos iPhone un certain nombre de messages publicitaires,

un rapport dressant un état des lieux de la fiscalité pesant sur les entreprises du secteur du commerce précisant les différences de prélèvement entre les entreprises du commerce physique et les entreprises du commerce en ligne, notamment transnationales.

des interfaces numériques permettant aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir en vue de la livraison de biens directement entre eux. Contrairement à la fourniture de services numériques, la vente de biens présente un degré élevé de substituabilité. L'utilisateur peut indifféremment obtenir le même bien auprès d'un utilisateur de l'interface numérique, d'un commerçant en ligne ou encore d'un commerce physique. termes, en ciblant spécifiquement le service de mise à disposition d'une interface numérique permettant la livraison de biens entre utilisateurs, la taxe sur les services numériques, dans sa mouture actuelle, aboutit à pénaliser les circuits courts de distribution par rapport aux circuits longs, dans lesquels vient s'interposer une grande enseigne entre le petit fournisseur et le consommateur final. Je le répète, le calibrage de la taxe et les nombreux effets d'incidence et de répercussion, souvent méconnus lorsque l'on crée une taxe, risquent finalement de renforcer les positions établies des quatre Gafa américains et d'envoyer au tapis les acteurs français et européens, soit l'exact inverse de l'objectif affiché.

et sur la désintermédiarisation destructrice de valeur, permise par certaines de ces plateformes. Quel est l'avis de la commission ?

En effet, les systèmes informatisés de réservation ne sont pas des interfaces mettant en contact les utilisateurs entre eux ; il s'agit d'un service proposant à ceux-ci un contenu numérique. La taxe sur certains services numériques n'a vocation qu'à appréhender les services dans lesquels ce sont les utilisateurs qui jouent un rôle déterminant dans la création de valeur. Or tel n'est pas le cas des systèmes informatisés de réservation, utilisés notamment dans le domaine des transporteurs aériens.

36 rectifié. La taxe sur les services numériques vise également à toucher les entreprises exerçant une activité économique sur un territoire où elles ne disposent d'aucune présence physique.

de se voir frapper par cette nouvelle taxe, ce qui aurait un impact non négligeable tant sur les capacités de recrutement du groupe que sur le secteur du voyage. Je précise en outre qu'il existe déjà un règlement européen qui encadre strictement l'utilisation des données SIR des voyagistes, empêchant de créer de la valeur à partir des données des utilisateurs. Les données SIR ne sont pas monnayées comme les informations recensées sur les réseaux sociaux qui enregistrent les données pour les revendre ensuite. Au regard de ces éléments, les SIR doivent être exemptés du champ de la taxe.

l'internaute qui la crée par ses recherches. Le Gouvernement devra préciser, notamment par instruction fiscale, le champ de la taxe pour éviter de taxer des activités qui,

La taxe sur les services numériques créée par ce projet de loi s'appliquera pour les plateformes proposant une multitude de services uniquement à la part de leur chiffre d'affaires résultant des sommes encaissées au titre de la fourniture des services taxables. Cet amendement vise donc à préciser le mode de calcul du montant de la taxe pour les entreprises proposant sur leur plateforme plusieurs types de services. Ainsi, tout abonnement payé dans le but de pouvoir accéder à un service de communication entre utilisateurs, sans que ses communications soient publiques, ne doit pas entrer dans le champ des activités taxables.

certaines entreprises, tout en fournissant une interface numérique, assurent également des services de logistique pour la livraison des biens. Ces services sont implantés sur notre territoire, fournissent des salariés,

possible, par un système de noria, de passer de l'un à l'autre. La mesure remet en cause le souhait du Gouvernement d'assurer une approche des offres multiservices qui soit pour la TSN cohérente avec l'approche retenue pour la TVA. Si elle était adoptée, cette mesure déboucherait sur un cadre juridique complexe et peu lisible.

et du rapport de Joël Giraud à l'Assemblée nationale, vise à clarifier l'article 1 pour s'assurer que le numérateur de la proportion est calculé en fonction des seuls messages publicitaires affichés sur l'interface numérique lors de sa consultation par un utilisateur localisé en France, et non en fonction de l'ensemble des messages publicitaires placés sur cette interface dès lors que cette dernière a été consultée par un utilisateur localisé en France.

n° 65. Cet amendement a le même objet : il vise à clarifier la règle de territorialisation des services de publicité. Il tend à préciser que seuls sont pris en compte pour le calcul du coefficient de présence numérique les messages publicitaires ciblant des utilisateurs localisés en France

introduirait une distorsion dans le taux effectif d'imposition entre les entreprises selon leur taille, ce qui serait contraire à la jurisprudence de la Cour

Le secrétariat d'État chargé du numérique est assez sensible à l'idée d'épargner les jeunes pousses françaises afin de leur donner les capacités de se battre contre leurs rivales des autres pays. Si nous pouvons examiner ce sujet au cours de la navette parlementaire, nous le ferons.

concurrence équitable entre les entreprises traditionnelles et les entreprises numériques et permettrait une meilleure contribution à l'impôt de la part du secteur du numérique, qui a été jusqu'ici sous-imposé Une telle augmentation ne serait en aucun cas confiscatoire ou abusive dans la mesure où le montant de la taxe constituerait une charge déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises redevables de l'impôt en France. En relevant le taux de la taxe, on incite les entreprises du numérique à déclarer leurs bénéfices en France. Je rappelle que le Conseil d'État

ses résultats mondiaux. En revanche, le passage de 3 % à 4 % pour un acteur fortement exposé en France, souvent plus petit, et souvent français pour le dire franchement, peut, lui, avoir des conséquences assez dommageables sur sa pérennité.

donc pour objet de créer un taux dérogatoire progressif à la taxe sur les services numériques, dans le cas particulier des places de marché proposant la revente et la livraison de biens. que les donneurs d'ordres abondent une redevance en fonction de la volumétrie carbone du transport qu'ils ont commandé et appliquent ainsi le principe pollueur-payeur ». Ce dispositif peut paraître complexe, mais il s'inspire d'un décret existant et vise à inciter la plateforme à utiliser des solutions de transport plus écoresponsables. En effet, ce mécanisme de remontée d'informations sur le volume de carbone généré par un transport a été inventé du temps du Grenelle de l'environnement. Un décret

Dès lors, les entreprises donneuses d'ordre, ici les plateformes qui livrent des biens, feront une déclaration directe de leur volume d'émissions de carbone, ce qui permettra de de moduler la taxe sur le numérique. Ce dispositif incitera les entreprises donneuses d'ordre à avoir moins recours à des modes de livraison dits « express » ou « rapides » et à des camions ou à des véhicules utilitaires dont la capacité volumétrique n'est pas

Il vise à instaurer un taux de 5 % lorsque l'entreprise numérique propose des services de livraison dont les coûts totaux excèdent les recettes demandées au titre des frais de livraison

à contester l'assiette proposée, à l'heure du réchauffement climatique et des problématiques générées par les transports en flux express.

il convient de mettre en place un dispositif de sanctions suffisamment dissuasif pour éviter toute dissimulation ou manipulation de données de la part des entreprises redevables. En l'absence de modalités de sanctions assez fortes, il est permis de s'interroger sur les démarches qui seront entreprises en la matière par l'administration fiscale. En outre, les seuils de redevabilité existants garantissent de fait que les entreprises assujetties disposent d'une expertise suffisante pour pouvoir renseigner efficacement et exhaustivement l'administration, sans que cela entraîne pour elles des coûts de gestion exorbitants.

ou C3S. La TSN est déjà déductible de l'assiette de la C3S, comme toutes les taxes assimilées à des taxes sur le chiffre d'affaires. La rendre par ailleurs déductible du montant de C3S lui-même introduirait un traitement inéquitable par rapport aux autres taxes assises sur le chiffre d'affaires, conduisant à un avantage non justifié pour les futurs redevables de la TSN. Dès lors que la TSN vise certains services numériques, cette déductibilité s'apparenterait à un avantage sélectif accordé spécifiquement à ce secteur.

La possibilité de mener des coopérations renforcées est souvent évoquée par le Président de la République, par exemple pour l'Europe de la défense. Pourquoi ne pas le faire pour la fiscalité numérique ?

Nous sommes à peu près sûrs que ce n'est pas nécessaire. Certes, la taxe sur certains services numériques n'est applicable qu'aux entreprises dont le chiffre d'affaires se situe au-delà des seuils d'assujettissement, ce qui conduit à placer hors du champ de la taxe les entreprises dont le chiffre d'affaires se situe en deçà. Pour Pour autant, ce dispositif ne peut être qualifié d'aide d'État, dès lors que les différenciations introduites s'appliquent à des entreprises qui, au regard des objectifs de la taxe, ne se trouvent pas dans une situation factuelle et juridique comparable. Le Conseil d'État a confirmé cette analyse dans son avis sur le présent projet de loi, indiquant que les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe ne sont pas dans une situation objectivement comparable à celles qui en sont exclues en raison de leur taille, compte tenu du modèle économique spécifique sur lequel leur activité repose. Un arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 mai 2019 relatif à une taxe progressive sur le chiffre d'affaires vient par ailleurs conforter cette analyse.

européens, la France continuera donc à avoir un taux supérieur à la moyenne européenne, ce qui ne correspond pas à l'engagement du Président de la République. Ayons le courage de le reconnaître, l'harmonisation fiscale européenne n'est qu'une incantation

à peine plus d'un an après avoir adopté la trajectoire de baisse pour la durée de la mandature, le Gouvernement demande une énième contribution exceptionnelle aux grandes entreprises. Sont ici visées 765 entreprises qui réalisent plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui inclut également des entreprises de taille intermédiaire, dont on jure par ailleurs, la main sur le coeur, vouloir favoriser la croissance et l'expansion

L'exemple britannique l'a montré : les recettes au titre de l'impôt sur les sociétés ont augmenté à mesure que le taux baissait.

Le scrutin est ouvert.